suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Depuis le début de l'examen de ce texte, nous cherchons- et nous en avons trouvé, avec la contribution du rapporteur -des dispositifs permettant d'associer plus étroitement le Parlement à cet état d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire.

par les mêmes motivations pour déterminer le système que j'ai précédemment exposé à notre assemblée et qui permet au Parlement de voter, à intervalles réguliers, la prorogation éventuelle du régime de l'état d'urgence et, à l'intérieur de ce régime, l'utilisation de pouvoirs pouvant aller jusqu'à l'imposition

un contrôle resserré du Parlement, autant je trouve que, dans cette hypothèse, nous ne pourrions plus rien faire d'autre ici que de discuter, avant même d'avoir pu dresser le bilan des mesures prises,

d'un rapport scientifique est particulièrement créative, mais ne me semble pas comporter une dimension d'utilité pratique très grande.

le décret déclarant l'état d'urgence sanitaire est obligatoirement motivé et le Parlement est déjà informé sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence. L'article 50-1 de la Constitution permet en outre de procéder à une déclaration,

2, supprimé en commission, qui proroge jusqu'au 1 avril 2021 l'application du régime de transition défini par l'article 1. En effet, il est indispensable de disposer d'un régime intermédiaire en sortie d'état d'urgence sanitaire.

restreignant moins les libertés publiques que les mesures de confinement qu'il avait prises à l'origine. Ce régime étant inutile, je ne vois pas pourquoi on le ferait durer, sauf, peut-être,

nous réclamer la possibilité d'utiliser des pouvoirs spéciaux jusqu'au 1 avril prochain sans avoir à revenir devant le Parlement. Ce n'est pas concevable ! La parole est à Mme

plusieurs régimes successifs qui ont tous la particularité de ne pas respecter l'exercice des libertés publiques. Vous avez tellement hésité sur cette législation

Ce dispositif fonctionne : au 21 août dernier, l'ensemble des consulats du réseau aux États-Unis avaient reçu 552 demandes d'exemption. Sur ce total, 401 personnes ont bénéficié d'une exemption. Le taux de délivrance s'élève De son côté, la compagnie Air France nous fait savoir que plus de 90 % de ses voyageurs entre les États-Unis et la France sont en mesure de présenter les résultats d'un test RT-PCR à l'embarquement et que la plupart des autres disposent d'une exemption.

des masques. Nous considérons que l'obligation de porter un masque pour des raisons de santé publique, dans les collèges, les lycées et les universités, dans les transports, les lieux clos, les entreprises et l'espace public de nombreuses villes françaises, implique cette gratuité : c'est

relèvent d'une solidarité nationale qui, en ces temps, est on ne peut plus nécessaire. Enfin, depuis le 26 juin dernier, les personnes souhaitant réaliser un test peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2. Ces examens sont intégralement pris en charge

rectifié. J'associe à cet amendement, mon collègue Teva Rohfritsch. Dans le cas de la crise sanitaire du covid-19, plusieurs arrêtés ont été pris en application d'une loi de pays adoptée par la Polynésie française. Ce texte prévoit, notamment, des contraventions de quatrième classe en cas de non-respect de dispositions telles que l'absence de port du masque. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 850 du code de procédure pénale ne permet pas, pour ces contraventions, d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire. Cet amendement a donc un objet simple, de bon sens, mais indispensable : rendre applicable en Polynésie française la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions aux réglementations mises en oeuvre localement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Quel est l'avis de la commission ? Favorable.

et en lui conférant des pouvoirs législatifs et réglementaires exceptionnels. L'objectif a été clairement défini par le Président de la République : nous sommes en guerre contre la covid et ses conséquences.

d'appliquer strictement la loi et de reconduire systématiquement dans leur pays les étrangers qui, par leurs agissements, constituent une menace grave pour l'ordre public leur a demandé « de mettre systématiquement en oeuvre les procédures à même d'interrompre, dans les meilleurs délais, la présence de ces personnes sur notre territoire ».

de rendre ces tests obligatoires dans les centres de rétention ou quand ces personnes font l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière d'origine administrative ou judiciaire.

C'est factuel ! La CNIL, dans sa délibération du 10 septembre 2020, rappelle que l'efficacité du prélèvement de ces données personnelles n'est pas avérée et demande que des indicateurs soient mis en place pour évaluer le rôle de ces dispositions dans la gestion de la crise sanitaire. Elle nous invite à renforcer l'évaluation et le contrôle permanent des mécanismes de manipulation des données personnelles et, ainsi, d'en mesurer l'efficience avant de les prolonger. Or nous nous trouvons dans l'incapacité de le faire, car de nombreuses inconnues demeurent

Je reconnais que le Conseil d'État s'est dit favorable à la prolongation des systèmes d'information ; en revanche, vous avez pu observer comme moi que les acteurs chargés de la collecte et du traitement des données dénoncent des insuffisances manifestes.

Le directeur général de l'assurance maladie regrette d'ailleurs cette entrave. Autre exemple : l'étude des chaînes de contamination est peu réalisable ; si les agents de l'assurance maladie ont connaissance des circonstances dans lesquelles le patient zéro a potentiellement contaminé ses contacts,

a entendu le président du conseil scientifique indiquer qu'il faudrait 20 000 à 30 000 personnes pour qu'un tel dispositif fonctionne. Celui-ci n'a pas fonctionné, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens

déclare favorable à leur maintien et à la prolongation dans la durée de la conservation des données pseudonymisées. Dans son avis public du 10 septembre, la CNIL ne remet pas en cause l'utilité des systèmes d'information. Par ailleurs, la prolongation de la durée de conservation des seules données pseudonymisées dépourvues de toute information nominative et destinées à la veille épidémiologique et à la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation est aujourd'hui fondamentale, compte tenu de la situation

Certes, pour le moment, c'est un échec. On peut d'ailleurs constater qu'un certain nombre de choses auraient pu être mises en place plus rapidement pour accompagner les brigades sanitaires, en particulier pour que celles-ci ne perdent pas de temps

amendement de permettre aux professionnels de santé scolaire et de l'enseignement supérieur ainsi qu'à d'autres professionnels de santé, étudiants en santé, de participer aux missions de gestion de la crise sanitaire et d'accéder, à cette fin, aux systèmes d'information, dans un même souci de traçabilité. Quel est l'avis de la commission ? Favorable.

de mes collègues Savary et Imbert, qui en sont à l'origine. Cet amendement vise à permettre, à titre dérogatoire et pour toute la période de l'état d'urgence, aux infirmiers exerçant dans un pôle de santé, dans une maison de santé ou dans un centre de santé d'effectuer des actes de pratiques avancées tels que la prévention ou le dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale, des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Le coût supplémentaire de cette extension serait largement absorbé, puisque son activité permettrait de faire plusieurs économies : les médecins pourraient déléguer plusieurs tâches afin de se concentrer sur des activités à plus forte complexité et donc à plus forte valeur ajoutée ; le coût horaire d'un infirmier en pratiques avancées (IPA) étant plus faible que celui d'un médecin, tout acte transféré à l'IPA serait vecteur d'économie ; enfin, les coûts organisationnels diminueraient en conférant directement à l'IPA un rôle d'adressage. L'habilitation sera automatiquement levée à la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Depuis mars 2020, quatre protocoles de coopération spécifiques et applicables en structures collectives permettent des transferts d'activité entre médecins et infirmiers. Ils ont été autorisés par arrêté ministériel. Par conséquent, le cadre réglementaire permet déjà ce type de pratique pour les infirmiers

dans les centres de détention ou de rétention, qui laisse des dizaines de milliers de personnes à la merci du virus : pas de gel, pas de masques et impossibilité d'assurer une distanciation physique. Nous savons que les cas de contamination en milieu carcéral explosent. Au 1 juillet 2020, on comptait près de 60 000 détenus pour 188 établissements.

il est véritablement impossible de garantir la sécurité sanitaire des personnels et des détenus. Il en est de même s'agissant de l'absence de campagnes de dépistage en prison,

être informé des conditions sanitaires des personnes détenues dans les établissements privatifs de liberté dans le contexte de l'épidémie de covid. Ce qui vaut pour les personnes détenues vaut évidemment pour les personnels de l'administration

pas de distribution de bouteilles d'eau, dans lequel elles n'avaient pas accès au gel hydroalcoolique, parce qu'elles auraient pu le boire. Comment assurer

Je remercie les auteurs de ces amendements d'avoir soulevé une question très grave. Il me semble toutefois que nous aurions avantage à la traiter à l'occasion de l'examen des budgets du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur,

critique. Puisque le problème est grave, il ne sera pas traité par un rapport que l'administration rédigera laborieusement, que le ministre tamponnera et qui sera transmis, s'il parvient jusqu'à ce stade, par le Gouvernement au Parlement.

C'est la première fois que je ressens viscéralement ce besoin d'essayer d'alerter, même si je doute de l'intérêt que portera le grand public à ce qui se passe derrière ces murs épais. « Je rencontre des gosses qui n'ont pas de masques et qui, pour certains, se sentent, sinon en danger, au moins délaissés. Ce n'est pas la première fois, et pour beaucoup ce ne sera, hélas ! pas la dernière. « Je porte un masque quand je vais les voir, quand je traverse ces couloirs étroits, quand je dois parfois attendre que la grille suivante s'ouvre, pressée contre des dizaines de détenus qui attendent aussi pour passer. J'emporte avec moi des masques chirurgicaux pour eux, pour les entretiens éducatifs que je mène dans une petite cellule aménagée en bureau de fortune. « Au mois de juillet, certains d'entre eux s'étonnaient : " On a besoin d'un masque ? Pourquoi, il est revenu le virus ? " Naïveté de gosse. Parce que, Parce que, oui, ce sont des gosses, persuadés que, si les adultes ne se protègent pas, ne les protègent pas, c'est que le virus ne circule plus ... Je me suis entendue murmurer qu'il n'était jamais parti, ce virus. « Impuissante,

Je ne peux que partager ce qui vient d'être dit : la situation est absolument dramatique à la fois pour les personnels et pour les détenus. Ici, ce n'est pas souvent le bon moment, c'est rarement le bon texte, ce n'est pas toujours le bon amendement, mais, pour le coup, je vais voter l'amendement présenté par Mme Assassi, pour le principe.

parties. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires tient à exprimer ses craintes quant au déploiement massif d'un mode de gestion dématérialisé susceptible d'engendrer plusieurs atteintes à l'effectivité de la justice. des dysfonctionnements informatiques peuvent nuire à la qualité des débats. En outre, la dématérialisation ne permet pas pleinement d'assurer la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. La solennité des audiences est fortement réduite cadre de ces procédures par écran interposé. Surtout, l'oralité des débats et le rapport humain en sont profondément bouleversés. Lors de la première vague de l'épidémie, de nombreuses violations aux principes fondamentaux de la justice ont été dénoncées par la Cimade. Ainsi, l'association l'association a constaté le recours systématique aux vidéoaudiences pour statuer sur les mesures privatives de liberté des étrangers retenus en centre de rétention administrative. Nous craignons pour cette nouvelle vague le retour de cette justice

Les conditions de mise en oeuvre de la justice ne doivent pas se faire au détriment du respect des droits de la défense. J'ajoute qu'une attention particulière doit être portée aux mineurs et aux personnes détenues, qui ont déjà beaucoup souffert de ces procédures dématérialisées lors de la première vague.

le maintien de cette dérogation, établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales, paraît nécessaire. Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l'application de ces dérogations jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. La parole est à Mme Maryse Carrère, présenter l'amendement n° 27 rectifié. Le rebond de l'épidémie de covid nous impose de réduire rigoureusement les contacts et les réunions. Naturellement, ces restrictions doivent concerner aussi le fonctionnement des collectivités territoriales, afin que celles-ci participent à l'effort collectif pour endiguer l'épidémie, mais aussi afin de protéger la santé des personnels et des élus locaux. Toutefois, il n'est pas envisageable que ces restrictions viennent heurter la continuité de l'action publique, tout particulièrement au

aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats mixtes ouverts restreints de se réunir par visioconférence ou audioconférence. En effet, cette possibilité ne leur est pas clairement ouverte par la loi, en sorte que, dans certains cas, la tenue d'une réunion par visioconférence ou audioconférence ou audioconférence a pu être refusée par le représentant de l'État dans le département, ce qui a rendu difficile l'avancée des travaux. Alors que l'état d'urgence sanitaire se prolonge, il apparaît important pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales que ces syndicats ne soient pas empêchés de fonctionner et que les interprétations des préfets ne varient pas d'un département à un autre. Tel est le sens de cet amendement de clarification. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement Cet amendement pourrait être tout à fait judicieux, si la règle qui n'est pas claire empêchait le recours à la visioconférence ou à l'audioconférence dans ces syndicats mixtes. Il me semble que l'ambiguïté

par téléconférence, les syndicats mixtes dits fermés, régis par les articles du code général des collectivités territoriales correspondants, et les syndicats mixtes dits ouverts restreints.

après avis de l'instance de dialogue social compétente. Ces lignes directrices de gestion doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources ; elles fixent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Ce dernier aspect est particulièrement important, puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus compétentes en la matière à partir du 1 janvier Or la crise sanitaire et le confinement ont fait prendre un retard important à nombre de collectivités territoriales dans les négociations sociales nécessaires à la définition d'un tel document. plutôt que d'obliger les collectivités territoriales à passer outre à la négociation sociale ou à y consacrer un temps disproportionné alors qu'elles sont concentrées sur le maintien de la continuité du service public, public, nous proposons de laisser un court délai, de trois mois, pour finaliser correctement cette réforme importante. Les décisions prises sur la base de ces lignes directrices de gestion, à compter, donc, du 31 mars 2021, pourront être rétroactives en application de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui permettra de ne pas léser les fonctionnaires concernés par un avancement ou une promotion.

favorablement accueillie par la commission, sur les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours dans la fonction publique territoriale. En la matière aussi, la crise

territoriale. Ces lignes directrices doivent déterminer la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, qui définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein d'une collectivité territoriale ou d'un l'établissement public. Leur adoption est l'une des mesures structurantes de la loi de transformation de la fonction publique. Le dispositif en vigueur n'impose pas un niveau de précision particulier en ce qui concerne les enjeux et les objectifs à déterminer. Ainsi, une collectivité territoriale pourra, dans un premier temps, privilégier des lignes directrices généralistes, dans l'objectif de respecter les délais fixés par la loi. Dans un second temps,

devant les employeurs territoriaux et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, je ne puis être favorable au report de la date d'adoption des lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale.

amendement s'inscrit dans la continuité de la prorogation par la commission des lois du maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. En octobre, 1,1 million de salariés ont été placés en activité partielle

également déposé par le groupe socialiste. L'épidémie et les contraintes qui en sont résultées ont naturellement pesé sur les entreprises et, plus généralement, sur toutes les structures dotées ou non de la personnalité morale : associations, groupements, fédérations. Afin de faciliter la réunion de leurs organes de direction, une ordonnance du 25 mars 2020 a autorisé celles dont les statuts ne le prévoyaient pas à se réunir à huis clos, c'est-à-dire à distance en recourant à tous les systèmes d'information envisageables- je crois que nous les avons tous expérimentés

un excellent amendement du rapporteur dont je partage à la fois la philosophie et la lettre, la commission a introduit dans le projet de loi cet article 3 , qui prolonge cette faculté jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette rédaction

-, il faut prévoir l'hypothèse où l'état d'urgence cesserait avant le 30 avril 2021 sans que la période transitoire qui suivra soit achevée à cette date. Dans ce cas, certaines personnes morales de droit privé pourront avoir intérêt à continuer à se réunir à huis clos, alors même que la loi, d'après la rédaction actuelle, ne le leur permettra plus. Je pense notamment aux fédérations sportives concernées par les jeux Olympiques de 2021, dont l'article 1 du décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020 prévoit qu'elles ont jusqu'au 30 avril 2021 pour renouveler leurs instances dirigeantes. Rendons-leur service dès maintenant en prévoyant qu'elles pourront, le cas échéant, le faire à huis clos, même après la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais pendant la période transitoire qui suivra. est l'objet de l'amendement n° 65. Par ailleurs, le code de commerce prévoit que les associations ou entreprises qui y sont soumises disposent d'un délai de six mois pour faire approuver par leur assemblée générale les comptes arrêtés au 31 décembre de l'année précédente- soit, pour les comptes arrêtés le 31 décembre 2019, jusqu'au 30 juin 2020. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-318 a différé ce délai de trois mois, permettant de ce fait à ces personnes morales de réunir leur assemblée générale jusqu'au 30 septembre dernier.

Je sais, monsieur le rapporteur, qu'on reproche souvent à la loi d'être bavarde. Mais si cela peut aider nos concitoyens, autorisons-nous-le

raison de la situation sanitaire. Si, au contraire, nous avons vaincu l'épidémie d'ici là et que le Gouvernement ne nous demande pas de prolonger les pouvoirs spéciaux, il n'y aura aucune raison de prolonger le dispositif de l'ordonnance au-delà

les entreprises en leur disant : allons-y une haie après l'autre, en prévoyant déjà ce régime jusqu'à

car le diable est dans les détails -est la question que vous posez sur la date limite d'approbation des comptes. Comme chacun le sait, une société anonyme, après avoir arrêté ses comptes, dispose d'un délai de six mois pour les faire approuver par son assemblée générale. Compte

de l'année suivante. Elle doit normalement faire approuver ses comptes par l'assemblée générale dans un délai de six mois suivant leur clôture, soit avant le 30 décembre. Grâce à l'ordonnance du 25 mars

Si elles savent qu'elles risquent de ne pas être remboursées, elles n'iront pas au spectacle, et tout le monde l'avis de la commission ? La commission a souhaité traiter de la même manière les voyages, les spectacles et les manifestations sportives. Le régime de l'avoir paraît approprié et ne lèse pas les consommateurs dans la mesure où, si l'on ne peut résoudre l'avoir par une consommation de voyage, de culture ou d'événement sportif au-delà d'un certain délai, il sera remboursé. Restons-en là, s'il vous plaît.

en cas de résiliation du contrat, un remboursement doit être effectif dans les quatorze jours si une autre prestation n'est pas acceptée par le client. Il y va de la protection du consommateur.

Dans le même temps, la maison mère, basée en Allemagne, a reçu 2 milliards d'euros de PGE, dont 100 millions d'euros uniquement pour la filiale française. Au lendemain du déconfinement, 600 des 900 salariés en France ont été virés

entreprises ont versé des dividendes ; huit ont même fait l'exploit d'augmenter leurs dividendes au cours de la période. Au total, 34 milliards d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires par les entreprises du CAC 40.

de la fin de cette autorisation administrative de licenciement : sa suppression était censée permettre de créer énormément d'emplois, mais ça n'a jamais été le cas. Je rappelle que nous discutons de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

la commission des lois. L'amendement n° 50, même s'il est inspiré par de bonnes intentions, me paraît largement contre-productif.

Imaginez qu'un salarié se trouve être le seul employé de l'entreprise-

elle se verrait interdire de le faire. On préfère donc dans ce cas que non seulement le salarié n'ait plus d'emplois, mais que l'artisan ou le commerçant n'en ait plus non plus et qu'il n'y ait pas de chance de redressement pour cette entreprise. Parfois les intentions les plus généreuses, surtout quand elles sont sur le compte d'autrui, peuvent se retourner

attention, d'autant plus que, quand on décide du versement des dividendes, parce que les comptes de l'année précédente ont été bons, la situation de l'entreprise, si la conjoncture s'est retournée, peut-être très mauvaise.

pour motif économique dans les entreprises dont les activités économiques ne sont pas affectées par les mesures de police administrative qui sont prises pour lutter contre le Vous observez pourtant que la frontière entre les entreprises qui sont affectées par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le covid et les entreprises qui ne seraient pas affectées- on se demande lesquelles

la situation actuelle ne permet pas d'envisager une interdiction générale et absolue de toute rupture des contrats de travail. Je connais- comme vous, je suppose -des entrepreneurs qui

Madame la ministre, mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à zéro heure trente, afin d'aller plus avant dans l'examen de ce texte.

Cet amendement vise à permettre la prolongation du nombre maximal de vacations pouvant être effectuées en 2021 dans la réserve civile de la police nationale. Il s'agit ainsi de renforcer les capacités opérationnelles des missions de sécurité intérieure de la police nationale pour faire face à l'épidémie de covid-19. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement inspire beaucoup de sympathie à la commission, parce qu'il reprend une disposition que nous avions

Je pense aux mesures relatives à la prolongation du dispositif d'activité partielle et du fonds de solidarité pour les entreprises en difficulté, à propos desquels le Premier ministre a fait des annonces importantes cet après-midi. Je pense également aux mesures relatives aux gardes d'enfants et à la continuité de l'accompagnement des personnes en situation de pauvreté. Ces mesures, dans un esprit partagé avec les mesures sanitaires décidées par ailleurs, ont une ambition cardinale : protéger les plus fragiles dans la période que nous vivons. Je pense enfin aux mesures permettant d'assouplir les modalités de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs organes délibérants ; elles sont de nature à garantir la continuité de l'action publique locale. Sur le fond, nous ne pouvons que soutenir ces dispositifs. Je pense que nous nous accordons tous sur ce point. Pour ce

nous ne pouvons nous en tenir à ce constat. Sur quoi nous prononçons-nous, alors que nous allons prochainement débattre d'un rétablissement de l'article 4 tel qu'adopté par l'Assemblée Nous débattons d'habilitations qui portent, à l'exception de deux d'entre elles- l'une a d'ailleurs été confirmée par notre commission -, sur des mesures que nous connaissons déjà : soit parce qu'elles ont été prises par de précédentes ordonnances auxquelles nous avions consenti, soit parce qu'elles ont été adoptées conformes dans la loi du 17 juin 2020.

L'exécutif ne s'est que trop livré à un exercice solitaire du pouvoir. Il est grand temps que le législateur retrouve sa pleine part dans le processus d'élaboration de la loi. Nous demandons donc la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? Vous de la commission ? Vous avez raison : légiférer par ordonnance dans la période actuelle est encore plus choquant que d'habitude. Par conséquent, il faut y regarder de très près. Précisément, si l'on regarde de très près, on fait un tri, tandis que votre amendement écarte toute possibilité d'accorder au Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnance. Or il y a des dispositions pour lesquelles nous pensons que c'est tout de même utile. C'est le cas pour l'aide aux entreprises, le chômage partiel, l'allongement des délais de paiement ou les règles de financement des hôpitaux, mais aussi pour l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Nous partageons le même souci de faire respecter les droits du Parlement. La demande du Gouvernement, qui portait sur 70 habilitations, était vraiment tout à fait excessive.

Je rejoins bien sûr l'avis du rapporteur sur certains points. Le Gouvernement considère indispensable de disposer d'une autorisation pour rétablir ou prolonger certaines mesures d'accompagnement

Madame la ministre, je vois que le Gouvernement n'est pas prêt à discuter avec le Sénat : il souhaite rétablir les 70 habilitations législatives. Pour autant,

vous rétablissez vos habilitations et vous ne tenez aucun compte de notre travail. Nous avons pourtant effectué un travail également très technique qui vous permettrait de trouver un accord avec le Sénat sur ce sujet essentiel. Comme vous êtes une parlementaire chevronnée, vous n'avez pas manqué de rappeler que vous partagez le souci qu'ont les parlementaires de ne pas déléguer le pouvoir législatif au Gouvernement sans raison impérieuse. J'ai compris que, compte tenu des délais très brefs que le Gouvernement a eus pour présenter son projet de loi, vous n'aviez pas eu le temps. Par précaution,

Ce n'est pas un petit fait ! Auparavant, lorsque vous placiez votre entreprise en liquidation judiciaire, ni vous, ni un ayant droit, ni un membre de votre famille jusqu'au second degré ne pouvait venir racheter partiellement ou totalement l'entreprise.

à supprimer des dérogations au droit du travail. Nous proposons de retirer deux dispositions maintenues dans le champ des habilitations qui vont être prolongées jusqu'en février et auxquelles nous étions opposés

l'avis de la commission ? Je voudrais dire à notre collègue Valérie Boyer que nous allons exactement dans la même direction : limiter drastiquement

de prévoir un certain nombre d'aides aux entreprises, telles que le chômage partiel, l'allongement des délais de paiement ou les règles de financement des hôpitaux ainsi que l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Je suis sûr que votre intention que ces mesures soient prises comme elles l'ont été, par ordonnances, dans la première partie de ce combat contre le

dans le secteur privé comme dans le secteur public. Je crois que vous avez raison de le souhaiter, puisque nous le souhaitons aussi. Une telle mesure devrait être débattue par le Parlement, après avoir été concertée avec les partenaires sociaux si elle était jugée opportune, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il en va de même pour les dérogations au droit du travail concernant les entreprises nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale exclu par le texte de la commission. Si vous acceptiez, vous aussi, de retirer les amendements n48 et 49, je crois qu'on gagnerait un peu de temps, puisqu'ils me paraissent tout à fait satisfaits. En revanche, votre amendement n°

2021. Nous ne pouvons affirmer que le covid sera toujours actif à cette période.

dernier : « Demain, les risques d'une seconde ou d'une troisième vague de covid-19 justifieront le maintien de ces dispositifs dérogatoires temporaires. »

que, par une simple ordonnance, on va mettre à bas ce qui fait l'intérêt et l'importance des conseils de surveillance des hôpitaux.

ensuite, prendre de telles mesures dérogatoires par rapport à leurs droits. La commission s'est livrée à un examen très approfondi de cette question. Elle en a conclu qu'il valait mieux laisser le Gouvernement prendre une ordonnance. Il ne s'agit que de dispositions budgétaires et comptables ; ce ne sont pas les piliers de la gestion de l'hôpital qui sont en cause. Si l'on devait attendre le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, on arriverait trop tard. Comme ce sont des matières essentiellement techniques qui n'appellent pas de grand débat de principe au Parlement, par exception à notre doctrine générale selon laquelle il ne faut pas accepter d'habilitation

il s'agit de permettre aux établissements de santé de se réorganiser et de concentrer l'ensemble de leurs moyens financiers et techniques sur la gestion opérationnelle de la crise, tout simplement. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie,

terme pudique -de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel. Nous voulons supprimer cette possibilité. Plusieurs d'entre

de la présence et de l'apport des médecins, de l'ensemble des personnels, des élus, de l'administration, des usagers. Vous ne pouvez Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'agit que de mesures financières. Ce n'est pas vrai ! Il faut regarder la vérité ! Nous sommes extrêmement attentifs à cette question, et c'est pourquoi nous tenons beaucoup à cet amendement.